rendement des DMTO, le gel d’une recette marquée par son dynamisme placerait plusieurs départements dans une situation proche de la cessation de paiements. Vu l’ampleur des investissements réalisés par les départements dans les services publics et les infrastructures, il est essentiel que les recettes de TVA affectées aux collectivités

de sérieux problèmes de mise en œuvre et d’équité, car de nombreux locaux sont imposables à la THRS alors même qu’ils ne constituent pas, à l’évidence, des résidences secondaires. Tel est le cas par exemple des salles de professeurs ou des maisons d’assistantes maternelles.

Nous proposons donc, dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités, soit respectivement les assujettis, les gestionnaires et les bénéficiaires de ces taxes, de fondre la TLV et la THLV dans la THRS, sans modifier les exonérations ni les zonages applicables.

comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

en matière d’hébergement d’urgence. Néanmoins, quelques aberrations compliquent la situation, notamment le fait que les propriétaires des logements concernés doivent parfois, alors même qu’ils font de l’hébergement d’urgence dans le cadre de l’intermédiation locative, payer

la fiscalité locale a été profondément réformée, notamment avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, je considère que le maintien de la liaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

de majorer la THRS ; les règles de liaison des taux. J’en viens, premièrement, à la fusion des deux taxes sur les logements vacants. Actuellement, vous le savez, la TLV est perçue par l’État et la THLV par les communes. avons déjà abordé ce sujet par le passé, et la position de la commission n’a pas changé : cette fusion, qui reviendrait à généraliser la TLV, mais en l’affectant aux communes, est une clarification souhaitable.

souhaitent qu’un logement meublé ne soit plus considéré comme un logement vacant. Deuxième sujet : de nombreux amendements tendent à exonérer tel ou tel type de local de la THRS.

de TFPB les locaux appartenant aux collectivités pour lesquels celles ci se paient la taxe à elles mêmes. Le troisième sujet a trait à l’extension de la faculté qu’ont les communes de majorer la THRS, soit en relevant le taux maximal de cette majoration, soit en élargissant le périmètre des communes éligibles. La commission, qui n’a pas souhaité augmenter la fiscalité pesant sur les contribuables, s’est opposée à l’ensemble de ces initiatives.

des règles de liaison des taux, selon l’expression utilisée dans le rapport du groupe de travail sur la décentralisation rédigé sous l’égide du président Larcher. cela signifie que la commission accepte la déliaison du seul taux de la THRS, à condition que son évolution reste encadrée.

envahis par les résidences secondaires. Dans une ville comme la mienne, on compte 7 000 résidences secondaires supplémentaires chaque année, et – il se trouve que c’est la ville la plus dense d’Europe – les possibilités d’y construire du logement neuf sont rares. Concrètement, les propriétaires occupants sont remplacés par des résidences secondaires, ce qui se traduit par une baisse de la population. Dès lors, la question est simple : nous donne t on la liberté de fixer les taux ? Nous ne demandons qu’une seule chose : laissez nous libres

est voté, il fait tomber tous ceux qui ont la même portée sur les mêmes éléments ou qui sont contradictoires avec lui. Cela étant, une discussion commune

sur la liste annexée au décret du 25 août 2023 peuvent majorer la THRS. Cependant, lorsqu’une commune nouvelle regroupe des communes dont certaines avaient institué la majoration de THRS,

pour 2024, le code général des impôts permet aux personnes domiciliées hors de France de bénéficier d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. Si cette disposition fut la bienvenue, elle ne constitue que l’ébauche du cadre légal réclamé de longue date par nos concitoyens établis hors de France pour le statut de résidence de repli. Le présent amendement de Yan Chantrel et du groupe SER vise à aller plus loin dans la création de ce statut, en permettant d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par

au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, peuvent parfois se justifier dans les zones où, comme à Paris, les loyers sont encadrés, mais ils doivent demeurer exceptionnels et ne pas participer à une inflation générale du coût des loyers pour les familles. Ils ont été prévus pour permettre d’aller au delà de l’encadrement des loyers au regard d’éventuelles caractéristiques exceptionnelles du logement et pour tenir compte de situations particulières. Mais cet outil est aujourd’hui utilisé pour contourner la loi. Notre amendement vise à prévenir ces abus, en taxant ces compléments de loyer pour inciter les propriétaires à revoir leur usage.

loi. J’en viens à cet amendement. L’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique a introduit l’obligation progressive pour les employeurs publics de financer une partie de la prestation sociale complémentaire couvrant les risques liés à la santé de leurs agents, afin d’aligner les conditions de protection sociale complémentaire du secteur public sur celles du secteur privé. Il est donc proposé, sur le modèle des contrats de groupe de prévoyance souscrits par les entreprises,

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les départements, et ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est affectée. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de porter à 20 %, au lieu de 18 % actuellement, pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra, en responsabilité, être compensée par les compagnies d’assurances. Enfin, il est important de rappeler que l’intervention décisive des sapeurs pompiers limite les dégâts et donc les dépenses des compagnies d’assurances. Il paraît donc juste que celles ci soient davantage contributrices au regard des besoins de financement des Sdis. En adoptant cet amendement,

monsieur le ministre, que le Gouvernement

le rapporteur général.

Le changement d’affectation serait neutre financièrement et sans incidence sur les moyens de la Cnaf, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de 1 milliard d’euros sur la branche famille pour l’année 2023. Les moyens des Sdis s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

de cet amendement ne fragiliserait pas le modèle financier de la Cnaf, qui est structurellement excédentaire et qui présente un solde positif de 400 millions d’euros en 2024.

Nous connaissons les effets de la suppression de la taxe d’habitation ; nous n’y reviendrons pas. Pour autant, il faut redonner aux maires le pouvoir et la mobilisation d’un levier d’autonomie financière par la mise en œuvre d’une contribution citoyenne financée par tous et fléchée uniquement vers la section d’investissement. Pourquoi cette section ? Je me contente de rappeler, monsieur le ministre, que le fonds vert est en nette diminution,

au financement des services

par la mise en œuvre d’une contribution citoyenne financée par tous et fléchée uniquement vers la section d’investissement. Pourquoi cette section ? Je me contente de rappeler, monsieur le ministre, que le fonds vert est en nette diminution,

Pour une commune de 500 habitants, cela représente une recette de 25 000 euros ; pour une commune de 6 000 habitants, de 300 000 euros ; pour une commune de 40 000 habitants, d’environ 1,25 million d’euros. Je le répète, cela ne coûte rien à l’État En résumé, cette contribution aux infrastructures communales permet de restaurer le lien entre le citoyen et l’élu, de maintenir l’investissement local et de soutenir l’économie locale.

Ce dispositif, introduit par amendement dans le projet de loi de finances pour 2024, visait à ajuster la fiscalité applicable aux éoliennes, leur permettant ainsi de bénéficier d’un régime d’exonération. Nous sommes évidemment

d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (Eespig) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.

est à M. Bernard Buis. Cet amendement de notre collègue Nadège Havet vise à autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent – si et seulement si elles le souhaitent – à exonérer de taxe foncière et de CFE les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils permettent d’alimenter l’équivalent de 1 000 logements.

Cependant, afin de répondre à la crise du logement tout en maintenant l’objectif du ZAN, cette possibilité serait circonscrite aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols. Quel

n° I 1000. L’article 1388 du code général des impôts prévoit que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif appartenant à un bailleur social peut faire l’objet d’un abattement de 30 % au titre des années 2025 à 2030 lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cet abattement est conditionné à la signature par l’organisme d’un contrat de ville et d’une convention, annexée audit contrat et conclue avec la commune, l’établissement public

Il s’agit donc de donner la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre une délibération pour appliquer un abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les ménages sous plafond de ressources, évidemment – qui acquièrent un bâti existant dégradé dont le coût des travaux de rénovation est supérieur à la valeur du bien, dans des conditions à définir par décret. Cette mesure favoriserait la mise en œuvre du zéro artificialisation nette,

qu’en fonction du risque observé.

Ce même article exonère de cette contribution les exportateurs des eaux minérales, dès lors que les livraisons ou transports de ces eaux se font en dehors du territoire national. des communes françaises voient les eaux minérales issues de sources situées sur leur territoire quitter la France sans que la moindre contribution soit versée aux communes et sans que l’eau soit, même pour partie, distribuée aux habitants. L’adoption de cet amendement aurait aussi pour effet d’instaurer un principe d’égalité entre toutes

entre les départements concernés se ferait au prorata de la valeur des biens situés sur leur territoire, afin de garantir une attribution proportionnelle du produit de la taxe en cas d’implication de plusieurs départements dans une même transaction.

Les modalités de cette taxe seraient particulièrement complexes, car son produit serait réparti entre les départements au prorata de la localisation des biens inscrits à l’actif des sociétés qui devraient s’en

le système des permet à certaines sociétés à prépondérance immobilière d’échapper à la cession de biens immobiliers inscrits à leur actif, privant les communes

mais entre 20 % et 30 % avant péréquation ! Or leur chute est abyssale, et en la matière la bataille des chiffres est lancée. En moyenne, ils auraient globalement chuté de 25 % en 2023.

je vous remercie

Cette taxe, qui est prélevée sur les personnes physiques ou morales dans les communes situées à moins de soixante minutes en voiture d’une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse, contrevient à notre sens au principe d’égalité devant l’impôt. En effet, elle entraîne des différences de traitement entre des contribuables placés dans des conditions semblables. outre, dans un contexte d’inflation et de difficultés économiques croissantes, nous estimons que le coût de ce projet ne doit pas reposer sur les entreprises et sur les ménages de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie.

que la taxe sur les friches commerciales ne soit pas intégrée dans l’assiette de la taxe spéciale d’équipement, il y a là un non sens ! Je mets aux

favorisant une égalité réelle entre communes rurales et urbaines. Quel

l’euro près le budget des communes, la loi de finances pour 2020 a prévu, à compter de 2021, l’institution d’un prélèvement ou d’un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous compensées.

En effet, en l’état, le coefficient correcteur appliqué aux communes nouvelles issues d’une fusion est figé au moment de la réforme ; il ne tient pas compte de l’évolution différenciée des bases foncières des communes préexistantes. Cela peut entraîner un prélèvement supérieur à l’addition de ce qu’auraient acquitté individuellement les communes concernées avant leur regroupement. Dès lors, celles ci peuvent se voir

cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen des projets de loi de finances 2023 et 2024.

sans préjudice du versement mobilité perçu, le cas échéant, par chaque AOM locale sur son ressort territorial. Le taux du versement mobilité peut être modulé à la baisse par la région en fonction de la densité de l’offre de mobilité et du potentiel fiscal de chaque EPCI, afin de tenir compte des spécificités locales. Le rendement d’une telle

modulé selon les projets locaux, une bonification étant possible après avis du comité régional des partenaires, garant d’une représentation équilibrée des acteurs du territoire. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, ces mesures visent à concilier l’équité entre territoires urbains et ruraux et le respect des recettes existantes des collectivités et de l’État. La parole

Express –, a été créée, dans la seule région Île de France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage,

imposent l’accélération de la décarbonation des mobilités, dans laquelle les réseaux de transport public, facilitant la mobilité du quotidien, ont toute leur place. Offrir d’autres solutions de mobilité à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence et d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées, tel est le défi à relever pour les AOM. Pour cela, ces dernières doivent poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité.

Maintenir une qualité de service optimale requiert la régénération des infrastructures existantes et la poursuite de leur développement. Or ces ambitions se traduisent par un mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les AOM.

un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins en matière ni de mobilités ni de gouvernance. En effet, elle comporte divers biais, entraînant inéquité et discontinuité territoriales. Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être. Sa complexité et son obsolescence deviennent, de fait, contre productives pour les raisons suivantes. D’abord, les notions issues de l’Insee ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir et n’ont aucun lien avec les préconisations figurant dans la LOM et avec la mise en œuvre des Serm. Ensuite, les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables. Elles créent de fait une discontinuité géographique au sein et

ainsi que celle des AOM. Il permet également de prélever le VMA à hauteur de 0,2 % dans les communes déjà au plafond du VM tout en maintenant la possibilité de prélever le VMA à son taux maximum, de 0,5 %, dans les communes n’ayant pas atteint le plafond.

en dehors du centre des agglomérations. Or les mobilités sont un sujet pour tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà sa modulation concertée et garantissent et garantissent une juste charge. Il paraît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices de la mobilité un pouvoir effectif de taux afin de garantir un financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des Serm, en pleine responsabilité pour les élus concernés. Le présent amendement vise ainsi à faire du VMA un levier réellement additionnel.

Cet amendement vise à supprimer le plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation de véhicules, actuellement fixé à 60 euros. Je sais que le rapporteur général fera un beau geste.

Cet amendement a pour objet d’étendre la latitude donnée aux régions de fixer les tarifs de la taxe sur l’immatriculation applicable aux véhicules en fonction de la source d’énergie de la motorisation.

à M. Stéphane Sautarel. La perception du produit de la mise aux enchères des quotas carbone dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission de l’UE, fortement dynamique, confère à l’État un espace budgétaire

la législation européenne que cette ressource soit fléchée, à hauteur de 50 % au moins, vers des actions tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et, plus largement, à faire face aux conséquences du changement

Par conséquent, il est proposé dans le présent amendement d’inscrire les autorités organisatrices de la mobilité comme nouveaux affectataires de la ressource. Les deux

ces baisses plus que prévisibles des recettes de l’État.

la rubrique des bâtiments exceptionnels ne relevant d’aucune catégorie d’habitation et de leur appliquer un taux théorique de rentabilité de 8 % de leur valeur vénale.

En effet, les monuments historiques sont plus souvent l’occasion de déficits que de profits. Aussi, cet amendement vise à poser le principe selon lequel l’évolution de la taxe foncière sur le bâti

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à lutter contre la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles, conformément à la loi du 14 novembre 2018. De nombreux acteurs publics et privés se sont engagés à réévaluer leur cahier des charges, mais – il faut bien le dire – aucun changement significatif dans les pratiques d’achat n’est pour l’instant six premières années de déploiement de ce programme, on a valorisé les acteurs vertueux, partagé des connaissances, signé de nombreux guides d’achat. Il semble aujourd’hui pertinent

pour conséquence une sélection plus durable de nos partenaires commerciaux et une valorisation des productions forestières et agricoles françaises. Le présent amendement

pour les compagnies d’assurances de plus de 500 salariés et à 0,5 % pour les compagnies d’assurances de moins de 500 salariés.

Cette indexation ferait progresser la dotation d’environ 491 millions d’euros, soit la somme nécessaire pour permettre aux départements d’assumer l’ensemble de leurs missions d’investissement et de redistribution.

les dépenses sociales explosent, avec notamment le financement du RSA, la protection de l’enfance, l’aide aux personnes âgées – autant de compétences transférées par l’État, mais dont les départements assument encore aujourd’hui 53 % des coûts. De l’autre, les recettes fiscales s’effondrent,

ce sont ces mêmes départements qui assurent les services publics de proximité indispensables à nos concitoyens. Ce sont eux qui agissent au quotidien pour accompagner les plus vulnérables, lutter contre les inégalités et garantir la cohésion sociale de notre territoire. Face à cette situation, notre amendement tend à abonder un fonds de sauvegarde à hauteur de 466 millions d’euros. déterminé selon les besoins exprimés par Départements de France, est indispensable pour soutenir les départements les plus fragiles. Laisser les départements s’effondrer,

Je veux remercier